ces véhicules plus légers consomment moins et peuvent être achetés par une grande partie de la population. La transition écologique doit reposer sur ces deux jambes : les incitations fiscales nous poussent à modifier nos achats et nos comportements, en contrepartie de dispositifs d’aide efficaces, accessibles au plus grand nombre, et qui réduisent à zéro le reste à charge pour nos concitoyens de la classe moyenne et les plus modestes. En ce sens, la transition écologique doit être synonyme d’amélioration des conditions de vie des Françaises et des Français,

En quinze ans, rappelons le, les SUV ont « vampirisé » le parc et accru l’insécurité pour les autres usagers en ville. Ils ont renchéri les coûts, entraîné des frais annuels supplémentaires à l’usage de plus de 400 euros et contribué, pour une part importante, à l’augmentation des émissions de CO2 du secteur des transports. Leur modèle économique, énergétique et environnemental

sont donc une aberration climatique à laquelle il nous faut répondre en créant, comme nous le proposons ici, une incitation à opter pour des véhicules plus légers. Le barème du malus écologique actuellement retenu demeure largement sous dimensionné, car il ne s’applique qu’à 12 % de véhicules vendus chaque année en France. L’abaissement du seuil à 1 500 kilogrammes dès 2026, que prévoit le Gouvernement dans ce projet de loi de finances, ne devrait rapporter que 150 millions d’euros de recettes supplémentaires dès 2025

les flottes professionnelles. La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a instauré le forfait mobilités durables (FMD), qui permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par les salariés qui se déplacent à vélo,

que l’objectif du forfait est d’encourager les salariés à utiliser des modes de transport plus propres et moins coûteux pour aller travailler, de nombreux freins à son déploiement persistent, empêchant une réelle prise en main du dispositif par les entreprises. Aussi, cet amendement vise à inclure les services de location

l’avis du Gouvernement.

aux véhicules de tourisme, des particuliers et des entreprises. Une telle mesure serait des plus pénalisantes en outre mer, car les particuliers sont généralement contraints de recourir à leur véhicule personnel, compte tenu de l’inexistence ou de la faiblesse des réseaux de transports en commun. D’une part, le coût prohibitif des véhicules en outre mer représente un obstacle à la modernisation de la flotte des particuliers. D’autre part, pour l’heure, les véhicules électriques ne sont

Nous ne pouvons ignorer le contexte particulier de la Guyane. La transition écologique, bien que nécessaire, s’y heurte à des réalités géographiques, économiques et infrastructurelles qui rendent le malus écologique difficilement applicable.

Cet amendement du groupe socialiste vise à créer une taxe sur les dépenses de publicité en faveur des véhicules polluants. Inspirée de la taxe sur certaines dépenses de publicité, cette nouvelle par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA, qui engage des dépenses concourant à la réalisation et la distribution de tout type de publicité – affiche, télévision, en faveur de véhicules polluants. Le seuil de pollution retenu correspond à celui qui figure dans la nouvelle réglementation européenne,

sa portée environnementale. Enfin, cette disposition accentue encore les inégalités territoriales en frappant plus durement les habitants des zones rurales et périurbaines. Pour ces raisons, je vous invite à supprimer cet article, qui ne répond ni à des exigences sociales ni à des objectifs écologiques.

Le présent amendement vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public

inspiré des propositions de la Convention citoyenne pour le climat et d’organisations de la société civile. L’idée est d’appliquer le principe pollueur payeur, en ciblant particulièrement les voyageurs bénéficiant de services haut de gamme et en préservant les passagers de classe économique. L’avion, mode de transport extrêmement polluant, bénéficie encore en France d’une fiscalité très favorable, notamment pour les jets privés.

un levier financier important pour accélérer la transition énergétique et moderniser les infrastructures ferroviaires, en soutenant la décarbonation du secteur des transports dans son ensemble.

que l’on ne nous oppose l’éventuelle inconstitutionnalité de notre dispositif, je rappelle que la politique fiscale entre dans le champ de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise les départements français d’outre mer à ne pas faire partie du territoire communautaire en matière de TVA. pour le tarif de solidarité sur les billets d’avion, la même dérogation doit pouvoir s’appliquer, dans les limites du respect des principes généraux du traité.

pour un montant qui devrait être compris entre 120 millions et 150 millions d’euros cette année. Dans le contexte budgétaire contraint actuel, chaque secteur doit naturellement prendre sa part au redressement des finances publiques. La hausse de la taxe est, en outre, la moins mauvaise des solutions, car elle est fondée sur la destination finale du passager ; elle limite donc les effets de distorsion de concurrence au profit des vols avec des escales hors de France. Toutefois, l’ampleur de la taxation envisagée par le Gouvernement, de surcroît sans étude d’impact, est trop massive.

des lignes d’aménagement du territoire, dont l’équilibre financier est actuellement garanti par le versement d’une subvention pour charge de service public, pourrait alors être complètement dégradé. Par ailleurs, le niveau de taxation sur l’aviation d’affaires commerciale, qui pourrait atteindre 3 000 euros par passager sur certains vols, est particulièrement élevé et menacerait la filière en France. C’est pourquoi le présent sous amendement tend à prévoir un doublement

Ce sous amendement tend à exclure l’application de l’augmentation de la taxe sur les vols aériens de la catégorie « Destination européenne ou assimilée

seraient très fortement affectés par le renchérissement des prix des billets d’avion. Par ailleurs, pour les natifs de ces territoires, qui font régulièrement des déplacements pour se rapprocher de leur famille ou par intérêt matériel et moral,

a pour objet de faire contribuer les passagers aériens à l’effort de rétablissement des comptes publics à hauteur de 1 milliard d’euros. Cet effort portera sur les trajets de l’aviation commerciale d’affaires – à hauteur de 150 millions d’euros et sur les trajets relevant d’un service aérien régulier – à hauteur de 850 millions d’euros – et passera par une hausse significative du tarif de solidarité prévu à l’article L. 422 20 du code des impositions sur les biens Or cette augmentation aurait pour effet de renchérir le prix des billets, dont le montant est déjà très élevé, sur ces destinations, ce qui se traduirait par une baisse de fréquentation de ces lignes et, par voie de conséquence, par une diminution de l’activité touristique,

En effet, la Corse, seule région à la fois métropolitaine et insulaire, dépend beaucoup plus du transport aérien que du transport maritime. En conséquence, la continuité territoriale dépend directement de l’accessibilité tarifaire du transport de voyageurs par voie aérienne.

par avion. Il convient donc, pour tenir compte des caractéristiques de ce territoire et de ses besoins de mobilité spécifiques, de maintenir le tarif de solidarité à son montant initial.

territoires. Nous estimons nécessaire de faciliter les liens entre l’Hexagone et les outre mer en mettant en place des navettes plus régulières, que ce soit pour les marchandises ou pour les habitants. Notre amendement vise donc à exclure de la hausse de la taxe de solidarité sur les billets d’avion les vols en provenance et à destination des outre mer. Dans un contexte où le coût de la vie y est déjà supérieur de 20 % à 40 % par rapport à la métropole,

de cette dernière. Au terme de la période en question, une évaluation sera menée par les services compétents pour analyser les conséquences économiques et sociales de la mesure. En effet, cette hausse n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact à ce jour, alors que celle ci, entièrement supportée par les compagnies aériennes, entraînerait inévitablement une augmentation du prix des billets pour les voyageurs.

de trois des quatre tarifs composant la taxe sur le transport aérien de passagers, à savoir le tarif de l’aviation civile, le tarif de solidarité et le tarif de sûreté et de sécurité.

comme le Gouvernement le sait et, en fait, comme tout le monde le sait, les voyages en jet privé sont un non sens écologique. Leur seule valeur ajoutée, à savoir gagner du temps, n’est même pas probante.

personnes qui voyagent en jet s’acquittent d’une compensation financière. Celle ci ne sera jamais à la hauteur des dégradations que nous paierons tous et toutes collectivement,

selon l’économiste Lucas Chancel, une personne faisant partie des 0,01 % des plus riches de la planète émet, quant à elle, 2 332 tonnes d’équivalent CO2 en Nos jet setteurs ne seront donc que fort peu dépourvus de ces quelques euros de justice environnementale versés à notre pays.

Merci

que cette mesure risque d’aggraver les inégalités entre la métropole et les outre mer, tout en accentuant la pression économique et sociale sur ces territoires. Il ne faudra pas s’étonner

par l’augmentation de la TSBA, on ne trouvera pas les moyens nécessaires, y compris pour sauver de petits aéroports d’équilibre du territoire, qui, taxe ou pas, sont en train de disparaître. Il vaut mieux un fonds